Monsieur le président,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

sous les réserves d'usage. Mes chers collègues, par lettre en date du 10 juillet 2019, le Gouvernement demande l'inscription à l'ordre du jour du mardi 23 juillet, après-midi, sous réserve de sa transmission, de la proposition de loi visant à faciliter la gestion et la sortie de l'indivision successorale et l'exploitation d'un aérodrome en Polynésie française, de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de transformation de la fonction publique. Le Gouvernement demande également l'inscription, sous réserve de leur dépôt, des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace et sur le projet de loi de règlement du budget pour 2018, ou de sa nouvelle lecture. Acte est donné de ces demandes. Pour la proposition de loi relative à la Polynésie française, nous pourrions fixer la durée de la discussion générale à quarante-cinq minutes et le délai limite pour le dépôt des amendements de séance au lundi 22 juillet, à douze heures. Pour le projet de loi de règlement, en cas de nouvelle lecture, nous pourrions fixer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance au début de la discussion générale. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Le Gouvernement demande également l'inscription à l'ordre du jour du mercredi 24 juillet des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles sous réserve de leur dépôt, des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi relatif à l'énergie et au climat et sur le projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport, ainsi que, sous réserve de sa transmission, de la deuxième lecture de la proposition de loi visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, initialement inscrite le jeudi 25 juillet. Acte est donné de cette demande. La durée de la discussion générale pour l'examen des conclusions des commissions mixtes paritaires sur la proposition de loi relative à l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles et sur le projet de loi relatif à la création de l'Agence nationale du sport pourrait être fixée à quarante-cinq minutes chacune. Nous pourrions fixer le délai limite pour le dépôt des amendements de séance sur la proposition de loi relative à l'organisation des communes nouvelles au mardi 23 juillet, à douze heures. Y a-t-il des observations ? Il en est ainsi décidé. Enfin, le Gouvernement demande le retrait de l'ordre du jour du jeudi 25 juillet de la proposition de loi visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie. En conséquence, le Sénat ne siégera pas ce jour-là.

inséré par le Sénat, visant à ce que le Gouvernement donne au Parlement les raisons de son refus de notifier la taxe sur les services numériques à la Commission européenne au titre des aides d'État.

texte initial du Gouvernement, dont l'objet était de revenir, en 2019, sur la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. Permettez-moi de prendre quelques instants pour évoquer cette mesure de pur rendement, qui constitue une contrepartie d'un certain nombre de dispositions prises pour répondre au mouvement des gilets jaunes.

le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement se condamnerait à ne pas pouvoir respecter son objectif d'atteindre un taux de 25 % en 2022, ce qui serait évidemment très dommageable pour notre compétitivité et la confiance des entreprises. Plus on repousse cet objectif, plus, par définition, il sera difficile à atteindre Le Sénat avait également adopté sans modification, dès la première lecture, l'article 1 prévoyant la remise d'un rapport. L'accord a dès lors été obtenu en commission mixte paritaire sans la manifestation d'aucune opposition, ce qui témoigne de l'important travail de compromis réalisé. À ce titre, je salue l'excellente collaboration avec mon avec mon collègue rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud. Dès la première lecture, les deux assemblées avaient validé le principe même de la création d'une taxe sur les services numériques reposant sur une assiette et des modalités qu'aucun amendement adopté ne tendait à remettre drastiquement en cause. En effet, nous partageons tous l'objectif d'assurer une juste répartition de l'imposition des entreprises, quels que soient leurs modèles d'activité, répartition qui tienne compte du développement du numérique. Or le système fiscal international actuel ne nous le permet pas. Une réforme est à l'étude, sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques, Elle pourrait se concrétiser plus rapidement que nous l'anticipions lorsque le projet de taxe avait été envisagé à l'échelon européen. Dans ces conditions, la solution dont nous discutons constitue

comme une étape temporaire, dans l'attente d'une décision multilatérale plus adaptée, que le Gouvernement espère aussi pousser au travers d'elle. Compte tenu de ces éléments, le Sénat avait souhaité

Juridiquement, la taxe sur les services numériques constitue un pari à bien des égards : son assiette vise à territorialiser des revenus générés par les utilisateurs français sans qu'ils soient effectivement déclarés en France, en s'extrayant des conventions fiscales internationales de répartition des bénéfices. Nous avons fait en sorte de sécuriser le dispositif, en réduisant les risques juridiques identifiés et les sources potentielles de contentieux. Peut-être, monsieur le ministre, reviendrez-vous sur les risques constitutionnels mixte paritaire est revenue sur l'exclusion du champ de la taxe des services par abonnement, ainsi que des systèmes informatisés de réservation.

le Sénat s'est préoccupé du risque de remise en cause de la taxe au titre des aides d'État. Sans préjuger le fond, il nous paraissait essentiel de respecter la forme, qui commande de notifier tout projet d'aide à la Commission européenne. Si la taxe était, par malheur, qualifiée d'aide d'État, sans notification préalable, elle serait invalidée quand bien même elle ne serait pas contraire aux traités européens.

je me félicite donc que la commission mixte paritaire ait conservé l'article 1 A : au moins, le Gouvernement devra justifier son choix auprès de la représentation nationale. Sur le dispositif de la taxe lui-même, il convient de noter que les initiatives du Sénat ont permis d'aboutir à deux compromis. Le premier permet d'exclure de l'assiette de la taxe les services connexes à la mise en relation des utilisateurs, dans des conditions économiquement fidèles à l'objectif. Cela concerne essentiellement la logistique. Le second aboutit à préciser les critères de localisation des terminaux en France, de manière à respecter les exigences de protection des données personnelles. Voilà l'accord auquel nous sommes parvenus. On peut toujours regretter que telle ou telle mesure ne soit pas retenue : c'est le principe même d'un compromis. mixte paritaire a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Désormais, la taxe sur les services numériques va pouvoir entrer en vigueur, concrétisant la volonté que nous avons tous de parvenir à une plus juste imposition des géants du numérique,

pour l'adoption définitive d'un projet de loi important, qui porte à la fois sur la révision de la trajectoire de l'impôt sur les sociétés et sur la taxation des géants du numérique. Je tiens à saluer

C'est une question de compétitivité vitale pour nos entreprises, qui doivent dégager des marges de manoeuvre pour investir, pour innover, pour connaître la réussite dans le combat technologique du XXI siècle.

deuxième sujet qui nous rassemble ce matin est la taxation des géants du numérique. Je veux rappeler que cette taxation n'est le fruit ni du hasard ni d'une quelconque lubie de certains États européens. Elle repose d'abord sur un diagnostic du nouveau modèle économique auquel nous sommes confrontés au XXI siècle. Aujourd'hui, la valeur est créée par les données, par leur accumulation, leur

Nous voulons construire, pour le XXI siècle, une fiscalité qui soit à la fois juste et efficace. Nous voulons imposer à ce nouveau modèle économique les mêmes règles fiscales que celles qui s'appliquent à toutes les autres activités économiques. C'est fondamentalement une question à la fois de justice et d'efficacité Comment pourrons-nous, demain, financer nos biens publics, nos investissements environnementaux, nos écoles, nos crèches, nos hôpitaux, nos collèges, si nous continuons à taxer ceux qui créent le moins de valeur sans taxer au même niveau ceux qui créent le plus de valeur, c'est-à-dire l'activité numérique et les données ? C'est donc un principe de justice et d'efficacité qui nous a guidés dans le combat que je mène depuis deux ans avec le Président de la République pour convaincre les États européens, un par un, d'avancer dans cette direction. La taxe que nous vous proposons ce matin a un taux de 3 %. Elle porte sur le chiffre d'affaires, qui est aujourd'hui la seule donnée disponible et crédible qui nous permette de mettre en place une telle

Je redis à cette tribune que, dès que l'OCDE aura adopté une solution crédible de taxation des activités du numérique, la France retirera sa taxe nationale. Je veux être très clair avec vous sur ce point.

Je me suis battu, depuis 2017, pour convaincre nos partenaires européens. Au début, nous étions deux pays, puis cinq, dès l'automne de 2017 : l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. À la fin du mois d'octobre, nous étions dix-neuf États.

Je ne me résigne pas à ce que, en Europe, une minorité puisse bloquer la majorité. Je considère que, s'il y a une conclusion à tirer de ces débats européens, bien la nécessité de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée pour les décisions portant sur certaines dispositions fiscales. Bien sûr ! Enfin, nous sommes face à une réaction américaine. Le représentant au commerce des États-Unis, M. Robert Lightizer, m'a écrit pour me signaler que l'administration américaine allait ouvrir une procédure au titre de la section 301 du de 1974 en raison de l'adoption de cette taxe sur les géants du numérique.

Je veux rappeler que c'est la première fois, dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la France, que l'administration américaine décide d'engager une procédure au titre de la section 301. Je crois profondément qu'entre alliés nous pouvons et nous devons régler nos différends autrement que par la menace.

plutôt que par des menaces ! Cela me semble de meilleure politique pour traiter cette question fondamentale de la taxation des géants du numérique. Très bien ! De manière plus générale, chacun voit bien que nous sommes aujourd'hui confrontés à l'émergence de géants économiques qui ont un caractère monopolistique. Ils veulent non seulement contrôler le plus de données créer de la valeur à partir de ces données, mais aussi aller plus loin encore, en échappant, faute de décisions, à un impôt juste et en mettant en place des instruments d'échange qui pourraient, demain, prendre la forme d'une monnaie souveraine. en tant qu'élus ou que représentants des pouvoirs publics, d'éviter l'émergence d'entreprises qui deviendraient des États privés et auraient tous les privilèges des États sans les contraintes et les contrôles qui vont avec. Ma détermination à mettre en oeuvre une juste taxation du numérique est donc totale, par souci de justice et par souci d'efficacité. Ma détermination, avec l'ensemble de nos partenaires européens, à instaurer un cadre de régulation des données qui protège la vie privée de nos concitoyens est elle aussi Ma détermination, enfin, à faire en sorte que le projet d'instrument d'échange mis en place par Facebook, dit Libra, ne devienne pas une monnaie souveraine qui pourrait concurrencer la monnaie des États est tout aussi totale, car je n'accepterai jamais que des entreprises deviennent des États privés ! La parole

ces paroles catastrophées furent prononcées par l'économiste libéral Paul Leroy-Beaulieu, en 1908, alors qu'était discutée l'une des premières initiatives parlementaires visant à établir, en France, un impôt sur le revenu.

J'ai souhaité entamer mon intervention par ces propos, car ils illustrent les débats, les exagérations, les craintes qui, souvent, accompagnent les projets structurants de certaines époques. À l'ère du capitalisme industriel et manufacturier, c'était l'impôt sur le revenu qui était au coeur des débats. Aujourd'hui, c'est le numérique qui prend toujours plus de place dans notre économie, qui modifie nos façons de produire et la répartition des richesses. Ainsi, en France, trois entreprises sur cinq sont passées au big data

Dans ce cadre, plus que le seul impôt sur le revenu, c'est la taxation des acteurs du numérique qui fait l'objet de toutes les controverses. Ces débats sont d'autant plus aigus que, d'une manière générale, l'imposition des sociétés tend à décroître.

Comme il y a un siècle, nous voyons clairement émerger la nécessité de rétablir la justice fiscale et l'efficacité économique. Hier, c'était l'imposition sur le revenu qui suscitait des cris d'orfraie ; aujourd'hui, c'est la nécessaire taxation des géants du numérique qui est la cible des critiques les plus acerbes. Hier, certains prophétisaient la disparition de toutes richesses ; aujourd'hui, d'autres pensent que tout un pan de l'activité économique est menacé. Mes chers collègues, il faut se rendre à l'évidence : nous n'en sommes,

taxe. C'est une bonne nouvelle, car une épée de Damoclès pesait sur cette taxe, pourtant bien maigre. Le rapport annuel que nous avions proposé est maintenu. Merci

Tout d'abord, cette taxe sur le chiffre d'affaires n'est pas un impôt sur les bénéfices des sociétés et ne répond donc pas à la logique d'un impôt intervenant après un cycle économique, applicable aux seules entreprises bénéficiaires. Nos interrogations portaient, et portent toujours, sur la capacité qu'auront les services fiscaux à vérifier les déclarations des bases fiscales imposables que les entreprises leur feront parvenir, mais aussi parvenir, mais aussi sur la répercussion de cette taxe sur les prix des publicités par les entreprises exerçant une situation de quasi-monopole. Enfin, il est bon de rappeler le contexte dans lequel ce texte nous a été présenté. Lors de la discussion générale au Sénat, nous avons montré que ce projet de loi répondait surtout

l'annulation des hausses de la fiscalité écologique- il s'agit là certes de répondre à une forte demande sociale ; pour autant, on n'a pas trouvé les moyens de financer la transition énergétique et les projets écologiques à hauteur des besoins

parvenue le 26 juin dernier à un accord sur un texte commun entre nos deux assemblées. Ce projet de loi est important, bien évidemment en termes d'équité fiscale et de recettes budgétaires, mais aussi pour l'image de la France. capable de jouer un rôle de pionnier en anticipant de futurs accords internationaux, que nous appelons de nos voeux. Il est encore capable de prendre des initiatives, l'absence d'un accord européen, « plombé » par la règle de l'unanimité, tout en s'affranchissant de la tutelle des États-Unis. Le président Trump lui-même, dans l'un de ces élans impérialistes qu'il affectionne, à moins que ce ne soit pour des raisons électorales liées à l'approche de l'élection présidentielle américaine, a demandé hier à son administration, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, une enquête sur l'instauration d'une taxe GAFA en France. France. J'ignore si le président Trump peut capter Public Sénat, mais sa marque d'intérêt pour le texte dont nous débattons ce matin est un réel honneur pour nous, même si elle n'est pas forcément inspirée par la plus grande bienveillance. Avant d'évoquer sur le fond la taxation des services numériques, dite taxe GAFA, je reviendrai sur l'article 2 modifiant la trajectoire de l'impôt sur les sociétés. Il convient en premier lieu de préciser, comme l'a fait le ministre en réitérant les engagements du Gouvernement et du Président de la République, qu'il s'agit non pas d'un changement de cap ou d'un reniement, mais simplement de différer l'application de cette mesure en 2019, peut-être en 2020, pour les seules grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Les TPE, PME et ETI bénéficieront bien, elles, de la baisse de l'impôt sur les sociétés, telle qu'elle avait été programmée. L'article 2 n'a pas été soumis à la commission mixte paritaire puisqu'il avait été adopté conforme par le Sénat

du moins inhabituelle. En effet, la commission de finances avait émis un avis favorable sur un amendement de suppression soutenu par le principal groupe de la majorité sénatoriale,

Si je fais ce rappel, c'est que, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joël Giraud, dont je partage l'analyse, « l'adoption conforme par le Sénat de l'article 2 sur le taux de l'IS a [ ...] rendu possible un accord sur le texte entre nos deux assemblées ou, à tout le moins, en a grandement accru les chances. Si je comprends bien, en ne suivant pas votre avis lors de l'examen en première lecture, monsieur le rapporteur, et celui de la commission des finances, nous avons rendu service ! En ce qui concerne la taxe sur les services numériques, les positions du Sénat et de l'Assemblée nationale n'étaient pas très éloignées. Les différences portaient plus sur les modalités, sur le périmètre et sur l'approche de la sécurité juridique. Je tiens à rendre hommage aux deux rapporteurs et aux membres de la commission mixte paritaire, qui ont validé cet accord sur un texte commun. Chacun a fait des efforts et des concessions, qui, à mon sens, n'affaiblissent pas la portée du dispositif mis en place, mais lui assurent sans doute un meilleur équilibre. Cette issue conclusive a été facilitée par le partage d'un objectif commun : assurer une plus juste répartition de l'imposition des entreprises, quels que soient les modèles d'activité. Il faut bien reconnaître que l'élaboration de mesures dans ce domaine n'est pas aisée et relève en partie de l'innovation. toutefois pas de manière totalement satisfaisante à tous les problèmes rencontrés, qu'il s'agisse de l'appréciation de la base de taxation, du risque de double imposition ou de requalification comme aide d'État pour les entreprises qui en seraient exonérées,

puisque le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée sont les deux notions comptables les plus proches, ce qui, économiquement, pouvait paraître assez logique. Cependant, à ce stade, il convenait avant tout de parvenir à un accord sur un texte commun, susceptible de servir de levier dans les négociations internationales, notamment dans le cadre des travaux de l'OCDE.

Si elle est évidemment un enjeu économique, l'adaptation de notre fiscalité au déploiement de l'économie numérique est aussi un enjeu éthique.

à peine plus de quatre mois après la présentation du projet de loi en conseil des ministres et après une première lecture ayant permis à chacune des deux assemblées d'enrichir et de consolider le texte initial. Je tiens à féliciter les deux rapporteurs, sans qui l'adoption d'un texte commun, renforcé, mais équilibré, n'aurait pu être possible. Sur les cinq articles que compte le texte final,

Je profite également du temps de parole qui m'est imparti pour saluer l'investissement de notre collègue Bernard Delcros, qui a eu l'honneur de représenter le groupe Union Centriste lors de la réunion de la commission mixte paritaire, mais qui ne peut malheureusement être présent aujourd'hui, car il est retenu dans le Cantal par l'accueil d'une mission parlementaire. Je ne reviendrai pas sur les limites, pour ne pas dire les imperfections économiques de la solution à laquelle nous parvenons à cet instant. Taxer le chiffre d'affaires, c'est en effet taxer aveuglément et sans distinction l'entreprise en pleine croissance qui n'enregistre aucun résultat et celle dont les résultats sont très élevés. Hélas, aucune technique de déduction n'était juridiquement admissible ni suffisamment solide au regard des règles fixées par les conventions fiscales internationales.

Il n'aura malheureusement pas prospéré, eu égard au risque d'incompatibilité qu'il présentait avec la réglementation européenne sur les aides d'État. La meilleure des solutions serait d'ailleurs peut-être, monsieur le ministre, de profiter de l'adoption de ce texte et de la création, même provisoire, de la taxe sur les services numériques pour supprimer la C3S, dont la nocivité a récemment été rappelée par le Conseil d'analyse économique. Quoi qu'il en soit, nous devons nous féliciter que bon nombre des modifications introduites par le Sénat à l'article 1 aient été conservées. Je pense à la clarification opportunément apportée sur la territorialisation en matière de publicité ciblée, au report d'un mois de la date limite de paiement de l'acompte en 2019, de celle de la fin de la période de référence retenue pour cet acompte et de la date limite pour opter pour le régime de groupe, ainsi qu'à l'importante précision introduite, sur l'initiative de notre rapporteur général, sur les modalités particulières prévues pour 2019.

Il est souhaitable en effet de réduire au minimum, et le plus en amont possible, les risques juridiques identifiés plutôt que de nourrir, en aval, lorsqu'il est souvent trop tard, un éventuel lourd contentieux, extrêmement coûteux et nécessairement préjudiciable pour notre pays et ses finances publiques. La remise par le Gouvernement d'un rapport sur les motifs de l'absence de notification de la taxe à la Commission européenne procède, dans ces conditions, de la sagesse la plus élémentaire. C'est là, on le sait, la marque de fabrique de notre assemblée Plusieurs modifications apportées par le Sénat ont par ailleurs fait l'objet de rédactions de compromis, qui nous satisfont parfaitement. Le souci que nous avons manifesté à travers le bornage temporel de la taxe, de la taxe, entre 2019 et 2021, a manifestement été partagé par nos collègues députés. La commission mixte paritaire a entendu les réserves que nous avons exprimées sur les fragilités d'ordre à la fois économique,

des utilisateurs, il tient compte de nos inquiétudes, s'agissant notamment de la protection des données personnelles, en retenant un dispositif qui s'inspire habilement de la rédaction de la proposition de directive de la Commission européenne du 21 mars 2018. un mot sur l'article 2, qui prévoit le report de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises en 2019, sur lequel les membres de mon groupe avaient porté en première lecture des appréciations diverses. À l'instar de Bernard Delcros, je considère cette mesure de rendement nécessaire et son adoption responsable, compte tenu des dispositions que nous avons adoptées en décembre dernier, alors que grandissait la grogne sociale d'un bout l'autre du territoire.

Sans doute imparfait, assurément insuffisant, ce premier pas demeure néanmoins décisif, car il permettra enfin de faire changer le système d'imposition applicable aux géants du numérique. Nul doute que la voix de la France sera une fois encore un accélérateur indispensable à l'émergence d'une solution internationale, quelles que soient les menaces du président Trump, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Nous voterons donc en faveur de ce texte sans réserve.

Ils ont permis d'apporter des améliorations substantielles au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale. Nous nous réjouissons également du succès de la commission mixte paritaire, qui démontre que l'ensemble des parlementaires sont conscients de la nécessité d'agir vite. texte est d'abord une question de justice fiscale, mais aussi une question de souveraineté, alors que l'Union européenne accuse un sérieux retard dans la course aux datas, richesses d'une nouvelle nature. À l'heure actuelle, la taxe sur les services numériques est la meilleure réponse que nous puissions apporter à la situation d'injustice fiscale dans laquelle se trouvent les entreprises qui opèrent en France. D'un côté, nos PME et nos ETI subissent les taux d'imposition les plus élevés de l'Union européenne ; de l'autre, de grandes entreprises internationalisées s'organisent pour ne pas acquitter en France

Mon groupe aurait ainsi préféré que cette nouvelle taxe porte sur le bénéfice, plutôt que sur le chiffre d'affaires, qui ne représente pas la capacité contributive des entreprises. Nous resterons donc vigilants à ce que cela ne se généralise pas à d'autres secteurs d'activité. En l'absence de consensus au sein des pays de l'Union européenne, la France fait aujourd'hui le choix de prendre les devants pour montrer l'exemple. Elle devra continuer à convaincre ses voisins de la suivre pour que le système se généralise à toute l'Union. Nous étions vingt-quatre États membres à voter en faveur d'un tel projet, mais il fallait l'unanimité

La nature multinationale des géants du numérique et la spécificité de leur modèle économique exigent une solution globale que seule la communauté internationale peut offrir. Nous nous réjouissons que la France assume ainsi ses responsabilités sur la scène internationale et ouvre la voie à une solution durable à l'échelle de l'OCDE. Nous espérons que nos partenaires suivront bientôt, afin d'aboutir le plus rapidement possible à la création d'une taxe globale sur les services numériques. Nous souhaitons de nouveau saluer les travaux de la commission des finances, qui ont également permis d'inscrire cette volonté dans le texte en intégrant une clause d'extinction. Celle-ci permettra de faire le point en temps utile. Plus que symbolique, cette taxe est cruciale dans un contexte où les géants du numérique s'imposent sans être imposés, tuant dans l'oeuf l'éclosion de nouvelles start-up innovantes. L'hégémonie économique est peut-être acceptée dans un pays qui y aspire, mais, en France, chacun paye son dû.

comme mon groupe le répète régulièrement, nous ne sommes ni dans l'opposition systématique ni dans l'adoption automatique. Au cas par cas, texte après texte, nous visons à conforter l'intérêt général, soit en adoptant les mesures qui vont dans le bon sens, soit en les modifiant. Concernant le texte dont nous discutons aujourd'hui, nous nous étions opposés en première lecture à l'article 2, qui reportait d'un an la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. Toutefois, cet article avait été adopté par le Sénat, malgré notre opposition. Par conséquent, la discussion en commission mixte paritaire portait essentiellement sur l'article 1, instaurant une taxation sur les services numériques. Cette taxe vise notamment les géants du numérique, surnommés les GAFA. Le 26 juin dernier, la CMP est parvenue à un accord sur ce sujet, chacune des parties ayant fait un pas vers l'autre, afin d'aboutir à un équilibre. Nous regrettons bien sûr qu'un certain nombre des mesures adoptées par le Sénat ne figurent pas dans le texte de cet accord. Je pense notamment à la limitation par le Sénat de la taxe aux seules années 2019, 2020 et 2021, cette dernière année étant la date envisagée pour parvenir à un accord au sein de l'OCDE. La majorité des députés a fait valoir que le bornage dans le temps de la taxe française pourrait réduire la pression mise sur l'OCDE pour aboutir à un accord international.

La majorité des députés a estimé que cette mesure aurait pu fragiliser juridiquement l'assiette de la taxe sur les services numériques. La disposition émanant du Sénat permettant aux redevables d'imputer le montant de la taxe qu'ils ont acquitté sur le montant de contribution sociale de solidarité sur les sociétés,

relative à la temporalité évoquée plus avant a été supprimée par la CMP, il a été expressément précisé, dans la partie demandant un rapport annuel au Gouvernement sur l'état d'avancement des négociations au sein de l'OCDE, qu'«

La volonté du Sénat de ne pas taxer un certain nombre de services logistiques ou connexes qui sont facturés aux entreprises sur les places de marché a été partagée par les députés ; une rédaction commune améliore et précise le dispositif. L'article 1 A, introduit par le Sénat, a été adopté conforme par la CMP, ce dont nous nous félicitons. Il prévoit que, en l'absence de notification préalable de la taxe sur les services numériques à la Commission européenne, le Gouvernement remet, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur les raisons pour lesquelles la taxe précitée n'a pas été notifiée à la Commission européenne. Cet article vise à mettre en garde le Gouvernement sur le risque juridique, lié à l'absence de notification transmise par l'exécutif à la Commission européenne, de remise en cause de la taxe au titre des aides d'État, la taxe ne visant que des entreprises au-dessus d'un certain seuil. Nous sommes ainsi parvenus à un texte plutôt équilibré. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains adoptera les conclusions de la commission mixte paritaire. La discussion

du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.